Monsieur le président, madame la Première ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, nos pensées volent vers l’Orient ensanglanté par les terroristes du Hamas, nourris par la haine, la barbarie et les actes génocidaires. Depuis 2007, la bande de Gaza est sous la coupe de ce mouvement islamiste qui veut détruire l’État d’Israël. Ses habitants subissent depuis le 7 octobre dernier, à la fois un blocus et des frappes qui font de nombreuses victimes civiles prisonnières des caciques du mouvement. Comment recréer l’espoir d’un monde meilleur chez toute une jeunesse palestinienne, rongée par la corruption d’une partie de ses élites et dont l’horizon se heurte aux murs de l’indifférence ? La solution à deux États, position exprimée avec constance par la France, paraît dépassée à l’époque où la Cisjordanie est devenue un immense gruyère du fait de la colonisation massive. À l’heure où le Président de la République veut non seulement soutenir la population et la démocratie israélienne traumatisée et fragilisée par une crise institutionnelle, mais aussi desserrer l’étau mortifère sur Gaza, des questions se posent. En particulier, l’idée d’une large coalition contre le Hamas interroge. De quelle nature serait elle ? Avec qui ? Avec quels moyens ? La constituer ne suppose t il pas d’intégrer le Hamas à la résolution déjà votée par les Nations unies contre l’État islamique ? L’ONU voterait elle cette résolution ? ? Surtout, comment une telle coalition pourrait elle protéger l’État d’Israël de ses voisins hostiles et éviter l’embrasement, pour créer à terme les conditions d’un retour à la paix ?

tous les otages, parmi lesquels on compte au moins une Française, est une priorité. Israël a bien évidemment le droit de se défendre face à un groupe terroriste qui a pour objet sa destruction. Dans le combat contre le terrorisme, les démocraties doivent être unies et solidaires, et c’est d’ailleurs pour cette raison que le Président de la République a évoqué l’idée d’une coalition

pour la réplique. Monsieur le ministre, sans réponse claire à ces questions, l’écho des pleurs et des lamentations hantera longtemps nos consciences. Il est urgent d’agir.

Territoires. Monsieur le ministre Clément Beaune, resterez vous sourd aux appels à arrêter le projet d’autoroute A69 entre Toulouse et Castres ? Vous annoncez depuis des mois que plusieurs projets routiers seront arrêtés parce que, à l’heure de la planification écologique, on ne peut plus faire comme avant : c’est vous qui le dites, et vous avez raison Alors, comment pouvez vous refuser de remettre en cause l’A69, ce projet autoroutier daté, typique d’un temps révolu où étaient clairement sous estimés les enjeux écologiques ? Votre ministère délégué est rattaché à celui de la transition écologique, pour lequel le Conseil national de la protection de la nature est chargé de l’expertise sur la biodiversité. Or ce dernier a émis un avis défavorable sur ce projet autoroutier. L’autorité environnementale compétente pour ce projet a aussi rendu son avis : elle a jugé ce projet anachronique, car reposant sur des données obsolètes. Par ailleurs, 1 500 scientifiques, certains comptant parmi les plus respectés à l’échelle internationale sur le climat, vous disent que l’A69 est l’un de ces projets auxquels il faut renoncer. Monsieur le ministre, que vous faut il de

il y a la légitimité d’élus qui ont porté ce vieux projet depuis longtemps. Bien sûr, il y a l’État de droit. Mais il y a aussi l’état d’urgence pour le climat et la biodiversité, la légitimité des générations futures.

Madame la ministre, les maires et les élus locaux expriment de plus en plus un sentiment de lassitude, voire de désespoir, avec pour corollaire un nombre important de démissions.

Face à la hausse de la sinistralité, les primes d’assurances et les cotisations flambent. En Meurthe et Moselle, Laxou, commune de 15 000 habitants ayant souffert des émeutes de juin, reçoit, sans contact préalable, un courrier de résiliation pure et simple dès le 1 janvier 2024. Dans le Nord, à Mont d’Halluin, un maire dont la commune est reconnue en état de catastrophe naturelle peine encore, des années plus tard, à obtenir réparation. Le maire d’Arcueil reçoit, bien que sa commune ne fasse pas partie des villes franciliennes les plus touchées par les émeutes, un avenant faisant passer de 1 500 euros à 2 millions d’euros la franchise à acquitter par la collectivité en cas de dommage Alors que les risques se multiplient – émeutes, saccages, inondations, retrait gonflement des argiles et autres risques climatiques –, des communes, notamment dans la Somme, se retrouvent démunies pour protéger leurs biens.

face au risque. En effet, sans assurance, elles ne peuvent bénéficier du régime de catastrophe naturelle. On imagine les conséquences financières en cas de sinistre grave… Face à cette situation, Madame la ministre, quelles mesures comptez vous prendre à l’avenir pour que toutes les collectivités puissent s’assurer ?

nombreuses collectivités rencontrent de plus en plus de difficultés à s’assurer, pour tout ou partie de leurs biens et de leurs activités. C’est un problème, surtout pour celles qui n’ont pas les moyens de s’autoassurer et de payer les dégâts en cas de sinistre.

Le sujet est complexe. Il est urgent, dans une première étape, de créer le dialogue. Nous avons obtenu en septembre la mise en place d’une médiation de l’assurance, qui est déjà à l’œuvre sur certains dossiers liés aux émeutes. Elle nous a permis, dans certains cas, comme celui de la commune de Mont Saint Martin où je me suis rendue la semaine dernière, d’obtenir le report de certaines résiliations et d’esquisser des solutions. Il nous faudra ensuite mettre des solutions sur la table, comme vous l’appelez de vos vœux.

réplique. Cette situation, difficilement acceptable par les maires, contribue à leur découragement dans l’exercice de leurs fonctions. Déjà, en 2019, notre collègue Sylviane Noël interrogeait le Gouvernement sur cet état de fait. Rien n’a évolué Les maires, notamment ceux des plus petites communes, attendent un réel soutien de l’État. Sinon, ils n’auront d’autre choix que d’abandonner. J’aurais pu citer d’autres communes ayant subi les mêmes constats de désassurance, comme Saint Brieuc ou Saint Omer. Ne leur restera t il qu’à se vouer aux saints pour se protéger ?

J’ai pu mesurer concrètement la semaine dernière, sur le terrain, les premières mesures que le Gouvernement a mises en place et qu’il faudra amplifier en 2024, car la crise est loin de se terminer.

En période de crise, on doit se serrer les coudes, loin des querelles de chapelle et des ego de chacun. Pour illustrer mon propos, je rappellerai que les élus de Mayotte, en sortant de leur rencontre avec le Président de la République vendredi dernier, lui ont adressé un courrier commun

Pouvez vous rassurer les collectivités locales, qui s’inquiètent de certaines rumeurs évoquant une reprise en main par l’État de leurs compétences dans le domaine de l’eau ?

devrons nous demander quel est le bon niveau de soutien et d’accompagnement de l’État aux collectivités territoriales. Merci pour votre engagement

Monsieur le ministre de l’agriculture, depuis début septembre, les cheptels bovins du Grand Sud Ouest sont atteints d’une maladie virale à forte contagiosité, la maladie hémorragique épizootique (MHE), transmise par un moucheron du type culicoïde. Les premières études engagées pour consolider nos données sur la mortalité de cette maladie fournissent des chiffres dans une fourchette allant de 0,3 % à 3 %. Nous notons également de nombreux avortements. Dans une majorité des cas, la guérison survient au bout de quelques jours, en traitant avec des anti inflammatoires non stéroïdiens très coûteux. Dans certains cheptels, plus de 50 % des animaux sont touchés. Les mesures de confinement mises en place dans un rayon de 150 kilomètres autour des foyers n’ont fait qu’aggraver les conséquences économiques de cette crise, puisque les éleveurs se sont vu interdire les marchés italien et espagnol. Depuis la mi octobre, ces marchés sont de nouveau autorisés, sous certaines conditions.

Quelles mesures prophylactiques pourraient elles être mises en place ? Le Gouvernement a t il prévu des mesures financières compensatoires afin d’aider les acteurs de cette filière bovine déjà rudement éprouvée ?

trop longtemps. Les cheptels diminuent et les éleveurs souffrent. C’est un nouveau coup dur pour ce fleuron de notre agriculture. Je compte sur le Gouvernement pour aider cette filière et nos éleveurs. La parole est à M.

C’est Véronique, 50 ans, qui vient de signer son contrat à durée indéterminée grâce au projet « territoires zéro chômeur de longue durée » au sein de l’entreprise à but d’emploi de Pontchâteau, en Loire Atlantique. Comme Véronique, plus de 3 600 personnes éloignées durablement de l’emploi ont pu retrouver toute leur place dans la société, mais surtout leur fierté et leur dignité.

L’Italie et la Belgique s’en sont inspirées, et le Comité européen des régions souhaite l’essaimer dans les pays de l’Union européenne. Or cette expérience est mise à mal par des choix budgétaires incompréhensibles.

malgré une augmentation apparente. Il manque 20 millions d’euros pour couvrir la baisse de la contribution au développement de l’emploi et accompagner les projets déjà engagés. Dans ce contexte, monsieur monsieur le ministre, quelles sont les mesures envisagées pour permettre le bon développement de ce projet exemplaire et pour faire en sorte que les 3 600 salariés de cette nouvelle entreprise ne soient pas condamnés à revenir à la case départ ?

La parole est à M. Michaël Weber, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

D’ailleurs, nos concitoyens ne s’y sont pas trompés : deux tiers des Français rejettent son utilisation. En 2017, la France a voté pour la première fois contre la réautorisation de cet herbicide dans l’Union européenne pour une durée de cinq ans. La voix de la France n’a cependant pas suffi pour obtenir l’interdiction européenne. Le Président de la République s’était à l’époque engagé à sortir la France du glyphosate « au plus tard dans trois ans », engagement qu’il a lui même enterré dès le fameux grand débat En 2019, les autorités publiques ont mis en place un plan d’action de sortie du glyphosate ; l’efficacité de ce plan s’est révélée malheureusement très relative. Voilà quelques jours, la France, par manque de courage, décide de s’abstenir lors du vote de la proposition de la Commission européenne sur le renouvellement de la licence d’utilisation du glyphosate pour dix ans dans l’Union il n’a manqué que deux voix pour obtenir son interdiction… Dans quelques jours, un nouveau scrutin devra définir la position européenne. Nous savons qu’en l’absence de majorité la Commission prendra la main sur la décision. Nous devinons, le cas échéant, quelle sera de l’agriculture, c’est une question de santé publique ! Quand comptez vous prendre vos responsabilités et sortir du double discours ? En définitive, quelle est la position de la France ? Depuis 2015, quels moyens avez vous mis en œuvre pour accompagner le monde agricole dans la recherche de moyens de substitution ? La

Monsieur le ministre, je crois surtout que vous n’êtes pas au rendez vous de l’histoire. Du courage, s’il vous plaît ! La parole est à M. Éric Bocquet, pour le groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

surtout, correspond aux profits que les grandes entreprises de la planète ont transférés vers les paradis fiscaux sur la seule année 2022, selon le bilan établi par l’Observatoire européen de la fiscalité rendu public lundi matin.

dans des pays comme l’Irlande ou les Pays Bas. N’est il pas temps pour le Gouvernement de mettre un terme décisif à cette concurrence fiscale dévastatrice et d’ouvrir enfin le chantier de l’harmonisation fiscale au sein de l’Union européenne ?

vous m’interrogez sur l’action du Gouvernement en matière de lutte contre la fraude. Je vais donc porter à votre connaissance les éléments transmis par le ministre délégué chargé des comptes publics, M. Thomas Cazenave, qui est retenu en ce moment même à l’Assemblée nationale et vous prie de l’en excuser. Le Gouvernement a présenté au printemps dernier, sur un sujet que vous connaissez bien, monsieur le sénateur Bocquet, un plan de lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques. Vous l’avez dit avec force : lutter contre la fraude, c’est d’abord, évidemment, s’assurer que chacun s’acquitte de sa contribution, mais c’est aussi un enjeu de cohésion sociale et un enjeu de finances publiques. Ce plan prévoit que 1 500 emplois supplémentaires soient consacrés directement à la lutte contre la fraude fiscale au sein même de la direction générale des finances publiques d’ici à 2027.

Nous avançons : les résultats du contrôle fiscal l’attestent. En 2022, ce sont près de 15 milliards d’euros d’impôts éludés qui ont été mis en recouvrement, un montant en hausse de plus de 25 % par rapport à 2018. La France est sauvée ! S’en féliciter, oui ; s’en satisfaire, non. Le Conseil d’évaluation des fraudes s’est réuni pour la première fois le 10 octobre dernier sous la présidence du ministre Cazenave. Il est composé d’une trentaine de membres, directeurs d’administration, experts internationaux, mais aussi parlementaires. À l’occasion de cette réunion, un programme de travail a été arrêté. L’objectif est de produire un rapport d’ici à l’été prochain. Encore ? Les représentants parlementaires ont été désignés par les présidents des commissions des finances et des affaires sociales de chaque chambre. complémentaires sont envisagées, comme la création d’un cadastre financier mondial ou la conduite de travaux pour une imposition minimale des particuliers les plus fortunés à l’échelle internationale. Dotés de ces nouveaux outils,

pour la réplique. Des paroles aux actes… Je crains, madame la ministre, que notre pays ne soit une partie du problème du fait des choix de votre majorité. En faisant adopter dernièrement, à l’Assemblée nationale,

La parole est à M. Michel Bonnus, pour le groupe Les Républicains.

sur le terrain et en dehors. Le sport n’a pas son pareil pour véhiculer des valeurs fortes, nobles, celles de l’effort, du travail, du respect, du collectif et de la solidarité. Le sport n’a pas son pareil pour cadrer des enfants, des adolescents, et en faire des adultes responsables, des citoyens attachés aux valeurs de la République. Nous ne remercierons jamais assez les éducateurs et les bénévoles de leur travail. Et je me réjouis que le Président de la République ait annoncé que le sport serait « grande cause nationale » en 2024. Le sport est un facteur d’émancipation et de liberté, j’en suis intimement convaincu… du moins en théorie. Car le sport, à l’image de notre société, est attaqué ! Pis, il est un des milieux privilégiés de déstabilisation de notre République et de promotion du séparatisme. Prière dans les vestiaires, port du voile sur les terrains, refus de la mixité, discours prosélyte antirépublicain, les attaques séparatistes se multiplient insidieusement, mais de plus en plus souvent ouvertement, au sein de nos structures sportives.

Les islamistes ne s’en cachent plus, d’ailleurs : les clubs de sport sont leur principale source de recrutement et d’embrigadement. Il y a quelques semaines, 69 clubs de basket ont conjointement réclamé la fin de l’interdiction du port du voile Gabriel Attal, ministre de l’éducation nationale, a fait preuve de fermeté et n’a pas tremblé en interdisant l’abaya dans nos écoles. Madame la ministre, ma question est simple, pour défendre les valeurs de la République il faut être ferme : êtes vous prête à interdire toute pratique dérogeant aux principes de laïcité et menaçant notre République ?

C’est en ce sens que j’ai fait diligenter au cours de cette année près de 3 500 contrôles de clubs sportifs, parmi lesquels 27, soit 0,8 %, ont donné lieu au repérage de signaux faibles de séparatisme. C’est toujours 0,8 % de trop, et il faut en effet prévenir les risques les risques là où ils se trouvent. D’où le plan d’action que j’ai mis en œuvre de manière résolue : 117 référents pour la prévention de la radicalisation déployés dans les services déconcentrés du ministère des sports, des référents citoyenneté mobilisés dans les fédérations, 6 000 contrôles

36 en 2024. Pour ce qui est du port du voile, j’ai salué la décision du Conseil d’État de valider l’article des statuts de la Fédération française de football indiquant que le port du voile pouvait être interdit en compétition pendant le temps et sur les lieux des matchs. J’ai conforté ce régime dans les statuts de la Fédération française de basket ball, et j’ai fait connaître à chacune des fédérations que dans l’exercice autonome de leur pouvoir réglementaire elles avaient la faculté d’ajuster leurs statuts pour coller à ces dispositions. Et le courage, en ce sens en leur donnant toutes les clés, y compris juridiques, sur ces sujets. Je le redis très fermement, ma main ne tremblera jamais pour faire utiliser les moyens que le Gouvernement a fait inscrire dans la loi en matière de contrôle du respect

La parole est à Mme Marion Canalès, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Aucun répit, aucun repli : aucun répit face à la crise sociale et au chômage, aucun repli pour cette expérimentation qui a déjà permis à 3 600 personnes de sortir de la privation d’emploi. Votée à deux reprises à l’unanimité par le Parlement, cette expérimentation a été saluée en 2020 par la ministre du travail de l’époque comme une « solution d’insertion sur mesure ». Elle a été coconstruite avec la société civile, et son utilité sociale et démocratique est citée en exemple par la Commission européenne ; l’Italie et la Belgique en dupliquent le modèle. À l’été, première saison, vous avez pourtant choisi de baisser la contribution de l’État au financement des emplois créés de près de 1 500 euros par an par À l’automne, deuxième saison, le budget prévisionnel, certes dynamique, se révèle ne pas être à la hauteur de l’enjeu : il est insuffisant. Il ne permettra pas la montée en puissance pourtant actée du dispositif, gèlera les perspectives d’embauche dans les territoires habilités et dans ceux qui sont prêts à l’être. Fragiliser le modèle, c’est précipiter l’échec. Pourtant, Pourtant, les résultats positifs sont visibles partout et dépassent largement le cadre de la personne concernée. En sept ans, à Thiers, dans le Puy de Dôme, le taux de réussite au brevet des collèges a grimpé de 12 %.

Les acteurs et employeurs privés et publics, ceux de l’économie sociale et solidaire, sont au rendez vous. Les effets positifs sont au rendez vous. Cela a certes un coût, mais cela n’a pas de prix ! De l’argent, il y en a, monsieur le ministre de l’argent, il en faut pour tenir les engagements pris : 20 millions d’euros. Quels moyens allez vous mobiliser durablement pour la France qui essaie, qui innove et qui fait la démonstration de sa réussite ?

95 % de prise en charge au niveau du Smic, c’est le plus haut taux de financement des emplois aidés connu dans notre pays. Toutes les structures d’insertion par l’activité économique aimeraient pouvoir bénéficier de la même chose ! Vous dites également qu’il faut accompagner tous les développements et toutes les perspectives.

Ma question s’adresse à M. le ministre de l’intérieur. La moitié des sénateurs de cette assemblée sort d’une campagne électorale, et le constat est très clair : les maires de nos communes rurales ont besoin de notre soutien pour se développer. Qui mieux que les élus pour connaître leur territoire et leurs besoins ? Qui mieux que les élus pour les soutenir ? Or, en septembre 2017, vous avez supprimé la dotation d’action parlementaire, dite réserve parlementaire, prétendument pour rétablir la confiance dans la vie politique.

surcroît, nous sommes particulièrement exigeants vis à vis des préfets quant à la façon dont la DETR est utilisée : elle doit aller partout, et elle va partout, y compris dans la ruralité la plus profonde. Vous le savez, les préfets consultent obligatoirement

administratif réalisé en chambre, mais dans un véritable dialogue avec les élus ; nous y sommes extrêmement attachés. Cette commission départementale réunit déjà de nombreux acteurs.

Notre démocratie demande que l’on renforce le lien entre le local et le national, entre le maire et le parlementaire, et que l’on redonne du pouvoir de décision aux élus nationaux dans un esprit de concertation

Le piège de cette nouvelle dépendance est en train de se refermer : vendredi dernier, le ministère du commerce chinois a annoncé qu’à partir du 1 décembre prochain il réclamerait un permis d’exportation pour certains produits en graphite. La Chine est le premier producteur de graphite du monde : elle assure près de 70 % de la production mondiale. Plus problématique encore, c’est elle qui raffine 90 % de la production planétaire de graphite.

d’août, la Chine avait restreint l’exportation de gallium et de germanium, métaux rares indispensables à la fabrication des circuits intégrés, des panneaux photovoltaïques ou de la fibre optique. Nous ne découvrons pas notre dépendance aux métaux rares chinois : l’Union européenne établit depuis 2011 une liste de matières premières critiques. En 2016, j’ai moi même rendu, avec Marie Christine Blandin, un rapport d’information pointant la nécessité de recycler les métaux des téléphones portables. En 2022, M. Philippe Varin a remis au Président de la République un rapport sur la sécurisation de l’approvisionnement en matières premières.

du graphite, qui est une matière première indispensable pour la fabrication de beaucoup de nos batteries, notamment pour la transition énergétique vers le véhicule électrique. Cette annonce fait suite à des décisions déjà rendues en juillet sur d’autres matières premières, comme le gallium et le germanium. Nous étudions l’impact de cette situation avec la délégation interministérielle aux approvisionnements en minerais et métaux stratégiques, et avec l’Observatoire français des ressources minérales

d’où l’intérêt des accords commerciaux et des accords internationaux que nous avons avec d’autres pays ou d’autres régions du monde pour sécuriser, précisément, les approvisionnements vers l’Europe.

dans le cadre des plans qui sont prévus à cet effet. Sous un Républicains. Ma question porte sur le soutien à la filière pêche, et j’associe ma collègue Vivette Lopez, sénatrice du Gard, à mes propos. Les pêcheurs vivent une crise sans précédent : aux conséquences du Brexit s’ajoute une envolée des coûts du carburant.

Même si toute l’enveloppe n’était pas destinée à la filière, il aurait peut être été pertinent d’augmenter les fonds consacrés à la pêche. En effet, de nombreux défis sont à relever. Il faut tout d’abord pérenniser l’aide aux carburants autrement que par des mesures d’urgence,

dont l’absence a des conséquences économiques importantes puisqu’il oblige les navires à faire un détour par Saint Malo ! La pêche est une richesse pour notre économie. Elle fait vivre nos littoraux au travers d’emplois non délocalisables et participe à la souveraineté alimentaire de notre pays.

Madame la Première ministre, le 10 octobre dernier, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté à une grande majorité un rapport ainsi qu’une résolution pointant de nombreuses violations par la France de ses obligations relatives à son adhésion au Conseil de l’Europe usage abusif du 49.3, surpopulation carcérale structurelle, problème avec la doctrine du maintien de l’ordre durant la crise des « gilets jaunes » et pendant les manifestations contre la réforme des retraites, questionnements sur l’indépendance de la justice, concentration des médias qui nuit au pluralisme… De plus, le 18 octobre dernier, le Conseil d’État s’est opposé à l’interdiction systématique des manifestations propalestiniennes, en contradiction avec une consigne du ministre de l’intérieur adressée aux préfets.

Ses travaux sont, sans conteste, d’excellente qualité. Néanmoins, vous n’êtes pas sans savoir qu’il s’agit d’une assemblée consultative, dont les rapporteurs choisissent eux mêmes le thème de leur rapport. Il n’est donc pas totalement impossible d’envisager que le choix de la thématique ait été guidé par quelques considérations politiques.

Madame la secrétaire d’État, vous vous dédouanez bien vite ! La France a également été condamnée à de multiples reprises par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) pour sa surpopulation carcérale

et qu’il était prêt à soutenir les propositions de la droite et des Républicains visant à s’asseoir sur nos obligations européennes, le tout après avoir attaqué la Ligue des droits de l’homme il y a quelques mois ! Il revient à sa famille ! Vous emmenez la France pas à pas vers un régime illibéral, et vous le savez

Il a démissionné, faute d’avoir été soutenu et protégé par les services de l’État, qu’il aurait pourtant alertés. En réponse à ces défaillances inacceptables, le Gouvernement a fait son, et et s’est engagé à travailler avec les élus pour assurer leur sécurité et prévenir les tensions, hélas ! prévisibles, notamment dans les projets d’installation d’hébergement d’urgence. Or le Gouvernement fait exactement l’inverse. Il vient de passer en force le 25 septembre dernier, contre l’avis unanime des élus locaux, le décret n° 2023 894 qui impose aux maires l’installation de centres d’hébergement d’urgence dans leur commune, sans leur demander leur avis et – cerise sur le gâteau ! – sans même avoir obligation de les en informer. Madame la secrétaire d’État, ne s’agit il pas d’hypocrisie d’État ?

le décret que vous évoquez pérennise un dispositif mis en place en juin 2021, qui a permis de faciliter et d’accélérer certaines opérations spécifiques et temporaires.

certaines constructions temporaires et démontables, telles que les résidences universitaires, les résidences sociales, les centres d’hébergement et de réinsertion sociale ou les structures d’hébergement d’urgence. d’urgence. Ce décret permet par exemple, dans une démarche d’urbanisme transitoire, de faciliter l’implantation de constructions temporaires destinées à l’hébergement d’urgence sur du foncier en attente d’urbanisation.

Ces opérations « à tiroirs », qui doivent rester exceptionnelles, peuvent se révéler incontournables pour la réalisation de certaines opérations de reconstruction du patrimoine social, de réhabilitation lourde ou de démolition dans le cadre de ces programmes. Ces règles ont donc été établies pour l’ensemble des structures d’hébergement, et non de manière spécifique pour les structures accueillant des demandeurs d’asile. La création de places d’accueil dans le dispositif national d’asile obéit à un schéma national décliné territorialement. Le Gouvernement a soutenu la création de 30 000 nouvelles places depuis 2017, ce qui démontre notre engagement à accueillir de manière digne les demandeurs d’asile. Pour organiser cet accueil dans les meilleures conditions, les préfets ont pour instruction claire du ministre de l’intérieur d’associer étroitement tous les élus à la création de nouvelles places d’accueil

Les représentants d’élus se sont prononcés à l’unanimité, et par deux fois, contre ce décret qui pérennise pour deux ans, et peut être plus, une situation prévue pour durer trois mois.

Vous le savez, ces derniers mois, les projets d’installation en Bretagne, dans la commune de Bruz, ou dans le Tarn, dans la commune de Réalmont, sont des échecs. En effet, en milieu rural, les services publics nécessaires à l’accompagnement, à l’éducation, à l’insertion et à la sécurité sont très insuffisants.

n’a pas de respect pour l’autorité locale, votre politique ne peut conduire qu’au désordre et à l’échec. La parole est à M. Damien Michallet, pour le groupe Les Républicains.

Comme tant d’autres élus locaux, je me suis retrouvé désarmé face à ces individus qui sont en réalité de fins connaisseurs de notre législation et qui ratent manifestement une brillante carrière de juriste… juriste… Dans cette situation, que fait l’élu local ? Il s’en remet à la justice ! Or force est de constater que si la saisine du juge aboutit – parfois – à l’expulsion des occupants illégaux, cette décision d’expulsion est rarement assortie d’une autorisation de recours à la force publique.

évacuation. Pourquoi ? Parce qu’en réalité l’ordonnance mentionne bien l’expulsion, mais l’autorisation du recours à la force publique est rayée d’un coup de crayon du magistrat… crayon du magistrat… Face à ces situations qui mettent à mal le moral de nos élus locaux, leur légitimité et parfois leur intégrité physique, pouvez vous nous éclairer sur la doctrine employée par le ministère de l’intérieur pour assurer l’application stricte des décisions d’expulsion ? en place tous les moyens nécessaires pour garantir aux élus que le recours à la justice, en France, n’est pas vain

des scrutins concernés. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels

âgées dépendantes (Ehpad) sont limités dans leur prescription aux résidents aux cas d’urgence et aux risques vitaux. Par ailleurs, on estime qu’environ un tiers des Ehpad ne disposent pas de médecin coordonnateur. Dans ces conditions, le suivi médical de leurs résidents peut s’avérer complexe. L’article 3 A, voté en première lecture à l’Assemblée nationale, vise à intégrer au sein des Ehpad le suivi médical des résidents. Toutefois, la rédaction adoptée rend le suivi médical par les médecins coordonnateurs obligatoire et garantit insuffisamment le respect du consentement des résidents.

Il ne faut pas faire de confusion entre le rôle du médecin coordonnateur, qui est maintenant chargé du suivi médical des résidents, et la fonction de médecin traitant. L’article 3 A permet de revaloriser le rôle du médecin coordonnateur dans les Ehpad en lui confiant explicitement la responsabilité du suivi médical des résidents.

De nombreuses tâches lui incombent déjà et sa responsabilité est renforcée par cette proposition de loi. Le problème de cet article – et c’est la raison pour laquelle la commission a supprimé deux alinéas –, ce sont les effets de bord.

comme l’indique l’exposé des motifs de cet amendement, le droit d’un résident à avoir un médecin traitant qui n’est pas le médecin coordonnateur, ce qui ménage une place à chacun.

pluriprofessionnelles (MSP) sont des outils majeurs pour l’accès aux soins de nos concitoyens. Face aux très grandes difficultés que connaît Mayotte en matière de démographie médicale, il est nécessaire d’apporter aux professionnels qui acceptent de se coordonner des possibilités assouplies et des garanties juridiques afin de favoriser la création de ces structures sur ce territoire spécifique. Cet amendement permet de créer une société interprofessionnelle de soins ambulatoires (Sisa) avec un seul médecin à Mayotte, ce qui facilitera la création de MSP et limitera les dissolutions subies à la suite du départ de médecins du territoire. La parole

Au contraire, la solution, adoptée par la commission lors de l’examen du texte, de supprimer la responsabilité illimitée et de consacrer une responsabilité limitée à deux fois le montant de l’apport constitue un alignement bienvenu sur les régimes les plus favorables au sein des sociétés civiles non immobilières. C’est une solution d’équilibre entre la protection des créanciers et la sécurisation des associés, qui permettra de lever certains freins à la constitution d’une Sisa. L’avis est donc défavorable. Quel est l’avis Gouvernement ? Madame la sénatrice, vous proposez de rétablir la responsabilité limitée des associés des Sisa au montant de leur apport dans la société, comme c’est le cas pour les souvent utilisées dans les cabinets médicaux de groupe. Rétablir la responsabilité des dettes des professionnels au montant de leur apport pour les Sisa s’approcherait donc de ce qui existe déjà pour les professions médicales exerçant en groupe. C’est en effet, comme le disait

besoin répété et durable de soins infirmiers. La restriction de l’infirmier référent aux seuls patients relevant d’une affection de longue durée (ALD) n’a pas de sens : le dispositif serait aussi utile à d’autres patients, tous ceux

tant sur l’amendement n° 196, qui permet à l’ensemble des patients de désigner un infirmier référent, que sur l’amendement n° 64, qui tend à faire de la désignation d’un infirmier référent une obligation pour l’assuré, et non plus une faculté. Plusieurs organisations représentatives des infirmiers nous ont indiqué qu’il était préférable de centrer la mesure, dans un premier temps, sur les patients ayant un besoin répété et durable de soins infirmiers.

la désignation universelle d’un professionnel de santé référent fait doublon avec la désignation d’un médecin traitant et crée une confusion. Il sera demandé aux patients de consulter en première intention l’infirmier référent, chargé de juger s’il est nécessaire de consulter un médecin, alors que ces deux professionnels ne font pas le même métier. Si la désignation d’un infirmier référent est subordonnée à la décision du médecin traitant

ne modifie pas la répartition des compétences entre professionnels de santé. Le médecin traitant demeurera le pivot de la prise en charge et du suivi des patients, comme de la coordination des soins. Toutefois, la désignation d’un infirmier référent peut s’avérer utile pour les patients souffrant d’une ALD et ayant fréquemment besoin de soins infirmiers

La désignation d’un référent doit relever de sa décision. Par ailleurs, les médecins traitants se plaignent déjà beaucoup de la surcharge administrative : une telle mesure ne ferait qu’ajouter une nouvelle gestion d’actes administratifs. Le médecin traitant doit évidemment être tenu informé de la désignation d’un infirmier référent par son patient,

La rapporteure a indiqué que les organisations infirmières ne souhaitaient pas une ouverture large du dispositif d’infirmier référent, ce qui est tout à fait juste. Elles nous ont dit la même chose, mais elles ont aussi

aujourd’hui, le volontariat de ces professionnels de santé ne permet pas d’assurer de manière effective la mission de service public de permanence des soins, au regard de la diminution continue du nombre de médecins volontaires. De ce fait, le soir ou le week end, les malades n’ont d’autre choix que d’appeler le 15 pour se rendre aux urgences, elles mêmes débordées. En cas de symptômes jugés insuffisants pour être pris en charge aux urgences, les malades se retrouvent sans aucune réponse médicale, si ce n’est

ça, c’était avant… Nous proposons donc – autre forme de gradation – que les négociations avec les organisations de médecins prévoient une revalorisation des tarifs sans reste à charge supplémentaire pour les patients, en contrepartie d’obligations de permanence

à la permanence des soins et consacre un principe de responsabilité collective. Nous reviendrons sur ce sujet lors de la discussion sur l’article 4 , qui concerne la permanence des soins ambulatoires ; je regrette que le présent amendement porte sur cet article… La commission a donc

La rédaction de l’article 4 concernant le « rééquilibrage » de la permanence des soins en établissement de santé issue des travaux de l’Assemblée nationale avait soulevé quelques préoccupations, que la commission a entendu prendre en compte. Ainsi, au delà des modifications apportées en commission la semaine dernière, le présent amendement vise à : préserver le schéma gradué que la commission a souhaité formuler, en insistant sur la responsabilité première des établissements ; assurer un fonctionnement opérationnel cohérent du présent dispositif et à permettre une participation active des professionnels libéraux, sans imposer de contrainte excessive d’exercice hors de leur établissement

L’article L. 1435 5 du code de la santé publique confie à l’agence régionale de santé territorialement compétente le soin d’organiser, avec les ordres professionnels concernés, la permanence des soins dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Une organisation efficace de la permanence des soins en établissements de santé ne peut être fondée que sur le volontariat. Par ailleurs, pour garantir la sécurité des soins, il est indispensable que les professionnels de santé participant à la permanence des soins en établissement de santé assurent cette permanence dans leur structure et aux côtés des équipes avec lesquelles ils travaillent habituellement. Pour ne pas déstabiliser cette organisation ainsi que celle des établissements de santé, la permanence des soins en établissement de santé doit donc s’effectuer dans le lieu habituel d’exercice des professionnels de santé volontaires. Cet amendement a été rédigé en concertation avec la Confédération nationale des unions régionales

La commission avait maintenu la notion d’appel à assurer la permanence des soins ou à y contribuer, adressé tant aux établissements qu’aux professionnels de santé. Le Gouvernement propose, pour sa part, celle d’invitation en cas de carence, ainsi que l’exercice d’une contrainte si la carence persiste.

enquête de la Cour des comptes à l’appui. Alors que le Gouvernement entend proposer un rééquilibrage de la permanence des soins entre public et privé, il nous a semblé peu opportun d’attribuer aux GHT une mission nouvelle en ce sens. Surtout, la commission a retenu un principe de réalité.

ou d’équipement matériel lourd à la participation de son titulaire à la permanence des soins, lorsque l’intérêt de la santé publique le justifie. Le directeur général de l’ARS arrête, dans le cadre du schéma régional de santé, un volet dédié à l’organisation de la permanence des soins qui fixe pour chaque zone d’implantation des objectifs en nombre d’implantations par spécialité médicale et par modalité d’organisation, avec un schéma cible du nombre de lignes de permanence des soins. Ce volet est opposable à l’ensemble des titulaires d’autorisations relatives aux activités de soins et aux équipements matériels lourds, ainsi qu’aux établissements et services qui viendraient à solliciter l’octroi de telles autorisations. 7 du code de la santé publique dispose que l’autorisation d’activité de soins peut « être subordonnée à l’engagement de mettre en œuvre des mesures de coopération favorisant l’utilisation commune de moyens et la permanence des soins répondant ainsi aux besoins spécifiques identifiés dans le schéma régional de santé. Selon nous, cette rédaction limite cependant le pouvoir contraignant du directeur général d’ARS aux dispositifs de coopération et mérite d’être clarifiée dans le cadre du meilleur partage de la permanence des soins entre les différents offreurs pour

de la commission ? Ces amendements identiques visent à renforcer le pouvoir de contrainte des directeurs généraux d’ARS la subordination de la délivrance d’autorisations d’activités de soins à l’effectivité de la participation à la permanence des soins.

pour les médecins régulateurs libéraux aux horaires de permanence des soins ambulatoires et en journée dans le cadre du SAS. Le présent amendement vise donc à étendre à l’ensemble des professionnels libéraux qui assurent la régulation des appels en permanence des soins et, en journée, dans le cadre

avaient réalisé au minimum une garde en 2020, selon le Conseil national de l’ordre des médecins. Autrement dit, le seul volontariat ne permet pas de garantir la permanence, donc la continuité des soins. C’est pourquoi cet amendement vise à faire en sorte que la participation à la permanence de soins soit partagée par l’ensemble des professionnels de santé.

La revalorisation du prix de la consultation n’a pas fait ses preuves, et l’engorgement des urgences est directement lié à un manque de gardes de la part de la médecine libérale.

L’article 4 ayant été supprimé en commission, nous souhaitons rétablir l’obligation à la permanence des soins en précisant qu’il est de la responsabilité collective des établissements de santé,

avec tous les professionnels de santé, notamment les médecins généralistes, pour dégager des créneaux, afin de répondre à ces demandes de rendez vous en journée pour des soins non programmés. Obliger

de l’internat est organisé à l’échelle nationale, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. Initialement, il était organisé dans sept interrégions, avant de l’être dans une zone sud et une zone nord, dont les contours étaient définis par arrêté ministériel. Il s’agit ici de rétablir une organisation par zones géographiques, ce qui permettra d’améliorer la démographie médicale et de lutter contre la désertification médicale.

et d’organisation du troisième cycle ont récemment été réformées, par un décret de 2016 et un décret de 2021. Il n’est pas souhaitable d’y revenir aussi tôt. La répartition des étudiants à l’échelon national lors de l’accès au troisième cycle permet de plus un meilleur appariement

C’est tout l’objet des politiques menées par le Gouvernement pour lutter contre les inégalités territoriales et sociales d’accès aux soins. Néanmoins, la régionalisation pourrait entraîner des disparités aussi bien dans la qualité de l’information délivrée que dans la répartition des professions de santé sur le territoire. Je mets aux voix

Attirer des étudiants dès leur formation, au moment de leur stage, constitue l’un des moyens d’y parvenir et de lutter contre les phénomènes de désertification médicale. L’article L. du code des collectivités territoriales, qui permet aux collectivités en zones sous denses d’attirer des aides aux transports et à l’hébergement, limite le bénéfice de ces aides aux seuls étudiants en médecine générale. Or les habitants des zones sous denses rencontrent également des difficultés d’accès à la médecine spécialisée. Il semble donc de bon sens et cohérent d’étendre cette faculté

aujourd’hui destinés aux étudiants en médecine et en odontologie, aux étudiants en orthophonie, afin que ces derniers puissent s’installer dans les territoires ruraux. Malgré un vote unanime de notre assemblée, le Gouvernement, en recourant à l’article 49.3, n’avait pas retenu cette proposition.

l’augmentation des moyens financiers et humains dans les universités de médecine n’a pas suffi à enrayer la baisse du nombre de professionnels formés. Selon la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), le nombre de médecins va continuer à baisser jusqu’en jusqu’en 2030. Le nombre d’étudiants inscrits en médecine est en dessous des besoins, de 20 % en médecine, 14 % en odontologie, 8 % en pharmacie et 4 % en maïeutique. Actuellement, les jeunes générations de médecins s’installent prioritairement dans leur territoire d’origine, proches d’un hôpital et de services publics de proximité. Notre amendement a pour objet de lutter contre les inégalités territoriales et sociales d’accès aux soins en définissant le nombre de places dans les formations de santé selon les besoins des territoires,

Il s’agit donc d’un dispositif hors internat, dont les modalités de mise en œuvre seront discutées avec toutes les parties prenantes, en particulier les organisations syndicales des étudiants de troisième cycle des études de médecine générale. notre proposition s’articule autour des départements. Les étudiants choisiraient leur futur lieu d’exercice sur une liste fixée par une commission départementale d’affectation et d’accompagnement.

de l’amendement n° 57 prônent la création d’une commission départementale d’affectation et d’accompagnement à l’exercice de l’année de professionnalisation qui serait chargée d’établir la liste des stages offerts aux étudiants en zones sous denses. La quatrième année du diplôme d’études spécialisées (DES) de médecine générale a été créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, qui a d’ores et déjà prévu que les stages seraient en priorité

Il n’est pas opportun de revenir sur de telles dispositions. Elles doivent s’appliquer pour la première fois en 2026 pour les étudiants qui se sont engagés dans cette spécialité en 2023.

vie. C’est le sens de la création de la quatrième année d’internat de médecine générale. Nous devons collectivement mobiliser tous les leviers disponibles. Nous avons d’ailleurs pris différentes mesures pour soutenir la réalisation de ces stages dans ces zones sous denses

prenons nos responsabilités pour apporter des réponses adaptées aux habitants de l’ensemble de nos territoires, afin qu’ils soient traités équitablement. Il y a urgence

Le scrutin est ouvert.

proches géographiquement d’une université dépendant d’une académie qui n’est pas celle de rattachement. Dans ce cas, les étudiants demandent des dérogations pour étudier au plus près de leur domicile, mais leur cursus ne les fait pas revenir sur leur territoire d’origine, où ils ont pourtant des attaches. Ainsi, les jeunes étudiants en médecine nivernais dépendent de la faculté de Dijon, mais demandent souvent des dérogations pour étudier à Clermont Ferrand ou à Tours. Ils sont issus d’un territoire terriblement sous doté qui a cruellement besoin d’eux. Pourtant, les stages, en particulier ceux de fin de cursus, ne leur sont pas ouverts. Dans le même temps, alors que la Nièvre dispose de nombreux maîtres de stage, les places de stage restent, pour beaucoup, non pourvues. En effet, les étudiants dijonnais rechignent à aller faire un stage dans la Nièvre, département le plus éloigné de la faculté. Il faudrait pouvoir proposer ces stages aux étudiants volontaires, là où ils se trouvent, et ce n’est pas forcément leur faculté de rattachement. Aussi, le présent amendement vise à permettre aux territoires qui ne sont pas dotés d’universités de proposer des stages aux étudiants où qu’ils soient. Toutes les études prouvent que les jeunes diplômés choisiront plus facilement de s’installer là où ils ont des attaches. Il est donc essentiel de leur permettre d’y faire leurs stages et d’y nouer des contacts au cours de leur cursus.

Toutefois, une telle modification bouleverserait profondément les modalités d’affectation des stages et soulèverait des difficultés opérationnelles : les stages sont aujourd’hui répartis, au début du troisième cycle, par ancienneté et selon le rang de classement ; ils le sont, en fin d’internat, par appariement des classements établis par les étudiants et par les maîtres de stage. Ces modalités de répartition sont difficilement envisageables à l’échelon national. Des dérogations sont d’ores et déjà possibles, permettant aux étudiants de réaliser des stages hors de leur région de rattachement.

La réglementation prévoit déjà la possibilité pour un étudiant de réaliser des stages hors de sa subdivision d’affectation, hors de sa région, dans les collectivités d’outre mer ou même,

faire passer les étudiants qui se destinent à être infirmiers par Parcoursup a été extrêmement délétère, au point qu’aujourd’hui, le taux d’abandon

L’expérimentation d’une orientation des lycéens issus de déserts médicaux vers les études de santé peut constituer un levier utile pour lutter contre la progression des déserts médicaux en France.

il est important d’encourager l’orientation des lycéens vers ce secteur. Actuellement, 50 000 postes sont à pourvoir dans les établissements et services des secteurs social, médico social et sanitaire, public et privé confondus. Si ces besoins ne sont pas nouveaux, ils tendent à s’amplifier : près de 150 000 postes seraient à pourvoir d’ici à 2025, soit près d’un quart des emplois actuels. De telles tensions touchent toutes les filières et toutes les professions. Elles s’observent particulièrement parmi les professionnels de l’accompagnement et du soin. Les métiers du soin et de l’accompagnement subissent des situations permanentes de sous effectif. En cause : un manque de reconnaissance des professionnels, la pénibilité du travail, des carrières trop peu attractives, des conditions de travail dégradées, mais aussi une crise de sens plus globale liée à la place accordée à ces métiers dans notre société. En amont, les formations spécialisées ne font plus le plein. Face à la pénurie de personnel dans les établissements médico sociaux et devant les difficultés de recrutement, il est important d’encourager l’orientation vers ces

d’être en réorientation en deuxième année si vous voulez entrer dans une formation de ce type. C’est complètement anormal ! Combien de jeunes sont refusés à la sortie du lycée dans les formations qui n’ont pas de capacités suffisantes ! Quel dommage face à la nécessité de former plus de soignantes et de soignants !

santé. Je crois en effet que c’est un levier extrêmement important. Pour le dire de manière très caricaturale, si les étudiants en médecine restent majoritairement des jeunes issus de familles CSP+,

Je ne suis pas sûre que cela suffise pour que vous acceptiez notre amendement, Madame la rapporteure, puisqu’il s’agit d’une demande de rapport, mais vous comprenez bien que c’est l’un des seuls moyens à notre disposition pour montrer la nécessité de réfléchir, de travailler à la création d’une année préparatoire aux études de médecine, précisément dans cet objectif de démocratisation. Nous savons que ces que ces premières années de médecine sont très difficiles et que beaucoup de familles font appel à des officines privées, parfois extrêmement coûteuses, pour passer ce cap. C’est en effet

Une année préparatoire post bac, avant l’admission au parcours accès santé spécifique (Pass) ne répond cependant pas aux objectifs de la réforme de l’accès aux études de santé. Celle ci permet aux étudiants ayant obtenu les 60 ECTS, mais non admis en filière à l’issue du Pass, de poursuivre en deuxième année de licence. Ainsi, les étudiants qui ont validé leur année universitaire, mais qui n’ont pas pu accéder à une filière de santé, poursuivent leur parcours et peuvent mobiliser une deuxième candidature au cours de leur cursus : c’est la fameuse licence accès santé (LAS). Créer une année dédiée de préparation sans débouché

est à Mme Silvana Silvani. L’alinéa 3 de l’article 6 prévoit que les groupements hospitaliers de territoire (GHT) pourront se doter de la personnalité morale dans des conditions qui ne sont pas détaillées ici ; elles seront définies par décret. Or, à la création des GHT, une telle possibilité a été repoussée pour éviter des déséquilibres territoriaux, et pour que la mutualisation de moyens au service des patients soit préservée.

La création d’une personne morale peut donner l’illusion d’une dynamique de coopération, mais elle ne résout en rien la question des moyens. Pour ces motifs, nous demandons la suppression de l’alinéa

À l’époque, le législateur considérait que la création et l’adhésion obligatoire à un GHT étaient une première étape suffisamment contraignante pour entraîner une recomposition de l’offre publique de soins. ont confirmé depuis toute leur utilité, notamment à l’occasion de la crise sanitaire, comme l’a relevé le rapport du Sénat sur la situation de l’hôpital et le système de santé en France du mois de mars 2022. Sept ans après leur création, il apparaît nécessaire de les doter d’outils complémentaires pour simplifier de nombreuses procédures et renforcer l’organisation territoriale des soins. L’article 6 de la proposition de loi crée ainsi un droit permettant d’opter pour la personnalité morale, pour ceux qui le souhaitent, afin de mieux répondre à leur mission.

propre des établissements parties de ces groupements, tout en ouvrant la voie à des simplifications majeures et à la mise en cohérence de certaines autorisations, aujourd’hui délivrées à l’échelle d’un établissement, pour des activités de soins

des personnalités morales des établissements avec la nouvelle, dont serait doté le GHT. J’avais d’ailleurs interrogé le Gouvernement sur sa vision de cette nouvelle personnalité morale, qui viendrait en quelque sort se superposer à celle des établissements parties quand elle ne résulte pas d’une fusion de ces derniers. C’est pourquoi nous avons inscrit dans le texte la semaine passée qu’un décret en Conseil d’État préciserait les conditions dans lesquelles un groupement hospitalier de territoire pourrait accéder à la personnalité morale, en prévoyant la demande conjointe de l’ensemble des établissements parties et le nécessaire accord du directeur général de l’agence régionale de santé, ainsi santé, ainsi que les modalités de conciliation des prérogatives respectives du groupement et des établissements parties. Une personnalité morale à statut particulier peut sembler une idée séduisante, mais d’une portée qui a semblé peu opérante à la commission. C’est pourquoi cette dernière n’a pas jugé cette option comme pouvant constituer une solution juridique solide. Par ailleurs, il n’est pas certain que la multiplication des statuts particuliers soit pertinente dans un paysage hospitalier déjà bien complexe.

Je vous en prie, la commission nous réunisse quelques minutes, afin que nous puissions étudier l’amendement de Mme la ministre et que celle ci puisse nous l’expliquer.